La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale

Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, comme je vous l'avais annoncé au mois de juillet dernier, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental Ce texte constitue la concrétisation de l'engagement du Président de la République de raviver le débat démocratique et d'accroître la participation citoyenne à l'action des pouvoirs publics. En effet, malgré les réformes successives qui ont élargi le champ de compétences du CESE, celui-ci n'a pas encore réussi à trouver la place qu'il mérite. Le Gouvernement entend remédier à cette situation avec un triple objectif : renforcer le rôle et la visibilité du CESE en sa qualité d'assemblée consultative, en faire un puissant levier de la démocratie participative, renouer avec sa vocation originelle de représenter les forces vives de la Nation. Je voudrais tout d'abord tenter de répondre à certaines de vos inquiétudes : il ne s'agit pas, et il n'a même jamais été envisagé, de faire du CESE une troisième chambre. Il ne s'agit pas non plus pour le CESE de représenter les collectivités territoriales, rôle que l'article 24 de la Constitution confère au Sénat. Le CESE demeure une assemblée consultative chargée d'éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre temps.

le CESE est largement sous-utilisé puisqu'il ne rend qu'entre 25 et 30 avis par an. Dans 80 % des cas, il le fait sur autosaisine. Pour y répondre, le projet qui vous est soumis développe principalement deux outils. D'abord, il renforce les liens du CESE avec les conseils consultatifs locaux.

Il faut mettre fin à ce cloisonnement et organiser des échanges fluides entre l'échelon national et les organes locaux, afin que le CESE puisse se nourrir des expériences et des connaissances territoriales. C'est l'objet de l'article 1 du projet de loi organique. Ensuite, le texte entend faire du CESE le carrefour des consultations publiques. Pour cela, il vous était proposé la création d'un nouvel article 6-1 dans l'ordonnance de 1958,

pour conserver notamment la consultation des autorités administratives indépendantes, celle des collectivités territoriales, ou encore celle des instances nationales dans lesquelles elles sont représentées. J'ai bien noté votre opposition à cette disposition et sa suppression par votre commission. Toutefois, et je ne fais que rappeler l'avis du Conseil d'État rendu sur ce texte, il s'agit d'une mesure de « simplification bienvenue et de nature à renforcer le rôle consultatif du CESE.

Pour redonner de l'attractivité au CESE, dont la qualité des avis est toujours saluée, le Gouvernement entend donc lui accorder une place prépondérante en matière de consultation. Vous craignez également un appauvrissement des études d'impact. Je crois que cette crainte est infondée. Avec le CESE, de regrouper au sein d'une même institution des profils et des compétences extrêmement variés qui seront pleinement de nature à assurer un avis d'une grande richesse, comme c'est d'ailleurs déjà le cas. Enfin, la discussion parlementaire à l'Assemblée nationale avait permis d'affiner le périmètre de l'effet substitutif de la consultation du CESE. Un bon équilibre avait ainsi été atteint, car environ la moitié des organes consultatifs ne seraient plus consultés en cas de saisine du CESE, tout en préservant la consultation d'instances éminentes, comme le Comité des finances locales (CFL). Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a déposé un amendement tendant à rétablir l'article 6 du projet de loi, dans sa rédaction issue de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale. Le deuxième objectif de la réforme renforcer la démocratie participative. Ce que nous voulons, c'est qu'à côté de la démocratie représentative, qui demeure le socle de notre fonctionnement démocratique, soit ajoutée une dose de démocratie participative, dans des proportions et un cadre maîtrisés. Pour cela, nous avions actionné deux leviers le recours aux pétitions ; l'organisation de consultations publiques et la participation directe de citoyens tirés au sort aux travaux du CESE. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à considérer que le droit de pétition est entouré de conditions de mise en oeuvre trop strictes, ce qui explique qu'il n'a jamais pu être exercé jusqu'à ce jour. C'est pourquoi le projet de loi prévoit trois modifications essentielles : d'abord, l'abaissement du seuil de recevabilité des pétitions de 500 000 à 150 000 signatures, pour qu'enfin cet outil de démocratie participative fonctionne ; ensuite, la dématérialisation des procédures, car il est temps que nous fassions entrer le droit de pétition dans le XXI siècle

voix au chapitre ? Ce serait une absurdité ! Ce progrès est non pas une concession faite à la jeunesse, mais un accélérateur de citoyenneté et une reconnaissance de ce qu'elle est capable de nous apporter : sa soif de débat. Le Gouvernement souhaite élargir le droit de pétition. Il n'est par conséquent pas question de l'assortir de nouvelles contraintes qui complexifieraient sa mise en oeuvre, comme l'institution d'une condition de domiciliation. En cela, nous sommes en désaccord total, madame la rapporteure -avec votre commission. Le projet de loi pérennise également l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat en consacrant l'organisation de consultations publiques, y compris par l'utilisation du tirage au sort, et prévoit la possibilité pour les citoyens tirés au sort de participer aux travaux du CESE. Lors de nos débats au mois de juillet dernier, j'ai bien noté votre opposition à cette pratique. Le président Retailleau l'avait d'ailleurs moquée comme un symbole de la « démocratie de la courte paille

Sans remonter à la démocratie athénienne, le tirage au sort existe dans de nombreuses démocraties, notamment à des fins consultatives : en Allemagne, en Irlande, en Islande, en Estonie, ou encore au Canada. En France, les jurés d'assises sont tirés au sort depuis la Révolution ! J'ai quelques raisons de penser qu'il faut défendre leur légitimité. Je précise, si besoin est, que le tirage au sort n'a pas vocation à supplanter le droit de vote. Il n'y a ni confusion ni concurrence entre, d'une part, l'intérêt de recueillir l'avis de citoyens tirés au sort et, d'autre part, l'exercice de la souveraineté nationale par les représentants de la Nation élus au suffrage universel. Mais renforcer la démocratie participative, ce n'est pas affaiblir la démocratie. Je crois au contraire que, plus nos concitoyens seront associés au débat public, plus la légitimité de ceux qu'ils éliront sera renforcée.